la première caractéristique du budget de la mission « Travail et emploi » en 2020, c'est sa stabilité par rapport à l'année précédente, stabilité faisant suite à plusieurs années de diminution des crédits. Les autorisations d'engagement se stabilisent cette année à 13,5 milliards d'euros, tandis que les crédits de paiement, portés à 12,8 milliards d'euros, connaissent une légère augmentation. La diminution des crédits de la mission constatée les années précédentes respecte strictement la programmation triennale 2018-2020 et traduit la nécessaire contribution du ministère du travail et de ses opérateurs au redressement des finances publiques. Cette trajectoire est également à replacer dans le cadre d'une amélioration de la situation de l'emploi. Selon l'Insee, au deuxième trimestre de 2019, le chômage, au sens du s'établit à 8,5 % de la population active, soit 0,6 point sous son niveau de 2015 et 2 points sous son niveau de 2015. Le chômage de longue durée- au moins un an -continue de baisser, s'établissant à 3,1 % de la population active, soit 0,4 point de moins qu'un an auparavant. La baisse constatée des effectifs du ministère s'inscrit dans le cadre plus large de la réforme de l'État et de son organisation territoriale. À l'inverse, les effectifs de Pôle emploi augmentent de près de 1 000 équivalents temps plein (ETP) en 2020. Cette évolution doit permettre un renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises. On sait les difficultés que certains chefs d'entreprise rencontrent pour recruter dans certains secteurs industriels en tension, comme la construction ou la métallurgie. Ce budget, comme je l'évoquais, s'adresse prioritairement aux publics les plus éloignés de l'emploi. Les parcours emploi compétences (PEC), lancés en 2018, constituent un progrès qualitatif certain par rapport aux anciennes formules de contrats aidés, qui visaient bien souvent davantage à améliorer artificiellement les statistiques du chômage qu'à répondre aux besoins réels et individuels des personnes. Les faibles performances de ces dispositifs en termes de sortie dans l'emploi durable sont là pour l'attester. Les acteurs du terrain semblent s'être emparés de la logique d'accompagnement renforcé qui avait présidé à la création des PEC. Peut également être relevé l'effort important en faveur du secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE), qui dépasse le milliard d'euros en 2020. Les structures de l'IAE accueillent les publics les plus éloignés de l'emploi, souvent peu qualifiés ou chômeurs de très longue durée. L'objectif est la création de 100 000 nouveaux postes dans ce secteur en 2022 par rapport à 2017, soit 230 000 personnes accompagnées. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et va donc au-delà de la politique de l'emploi. Le principal enjeu, maintenant, pour les structures de l'IAE est d'être en mesure d'absorber cette hausse de leurs moyens et de leurs effectifs. Le plan d'investissement dans les compétences (PIC) constitue un autre volet important de ce budget. Il se fixe pour objectif de former 1 million de jeunes décrocheurs et 1 million de chômeurs de longue durée, en mobilisant près de 14 milliards d'euros sur cinq ans. Une grande partie de sa mise en oeuvre relève des régions. Ces crédits seront en réalité diminués de 120 millions d'euros. Il était en effet nécessaire, pour préserver l'équilibre de ce budget, de compenser financièrement la suppression de l'article 79 du présent projet de loi de finances, suppression que nous approuvons. En effet, la mesure cet article, qui entendait restreindre le bénéfice des exonérations applicables aux aides à domicile, aurait ainsi pénalisé un grand nombre de nos concitoyens. L'impact de cette minoration de 120 millions d'euros sur le bon déroulement du PIC devra être évalué à l'aune d'une probable sous-consommation des crédits. Une difficulté qui ressort des auditions que nous avons conduites concerne également le pilotage du plan. On peut déplorer un déficit de coordination entre l'État et les régions. Il convient par ailleurs de s'interroger sur la pertinence d'un découplage des compétences d'accompagnement des jeunes, qui relèvent des missions locales, et des compétences de formation professionnelle, qui relèvent des régions. Dans l'ensemble, ce budget me paraît toutefois sérieux, en phase avec la situation de nos finances publiques et en phase avec les enjeux actuels de la politique de l'emploi. Sous réserve de l'adoption d'un amendement, que j'ai déposé avec ma collègue rapporteure spéciale Sophie Taillé-Polian et qui vise à renforcer les crédits consacrés aux maisons de l'emploi- comme l'année dernière et comme l'année précédente

L'amélioration apparente du taux de chômage ne saurait justifier une telle cure d'austérité pour le ministère du travail. Car les statistiques sont à prendre avec précaution. Force est de constater que certaines catégories d'actifs restent très éloignées de l'emploi. Je rappellerai quelques chiffres : le taux de chômage des jeunes s'établit à 19,2 % en 2019, soit 0,6 point de plus qu'un an plus tôt. Le taux de chômage des travailleurs handicapés s'élève également à 19 %. Ces évolutions s'inscrivent également dans un contexte d'augmentation constante des emplois précaires, qui est une tendance de fond du paysage social français liée aux politiques de flexibilisation du marché du travail.

à 83 % en 2017. La traduction la plus regrettable de ces orientations budgétaires est la baisse constante des effectifs du ministère du travail. Les emplois sous plafond ont diminué de près de 10 % depuis 2017, alors même que la situation de l'emploi, comme je viens de le démontrer, nécessite plus que jamais un renforcement de l'accompagnement et des moyens humains. Action publique 2022 » et « organisation territoriale de l'État » sont les autres noms de l'affaiblissement de la présence du ministère du travail sur le territoire. La hausse des effectifs de Pôle emploi cette année est louable en soi, mais celle-ci ne compense pas les réductions d'effectifs de ces deux dernières années. L'on ne saurait de surcroît attribuer le mérite de cette hausse au Gouvernement, car nous constatons cette année une nouvelle diminution, à hauteur de près de 10 %, de la subvention pour charges de service public de Pôle emploi. La hausse du nombre d'emplois à Pôle emploi est financée par une augmentation de 1 point de la contribution de l'Unédic, ainsi portée à 11 % de ses ressources. qui a par ailleurs imposé une réforme de l'assurance chômage restreignant considérablement les droits des demandeurs d'emploi dans le seul but de générer 4,5 milliards d'euros d'économies, fait ainsi supporter aux chômeurs eux-mêmes le coût du service public de l'emploi. C'est dans ce financement du service public de l'emploi et non dans une prétendue générosité excessive du système d'assurance chômage qu'il faut chercher la cause de la dette de l'Unédic. On peut également souligner la baisse très importante- ils ont presque été divisés par cinq -des moyens consacrés aux contrats aidés sur les dernières années. Cela a notamment un impact fort sur le tissu associatif, où ces personnes accomplissaient des missions diverses et très utiles socialement. J'aimerais revenir maintenant sur l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ». Je rappelle son fonctionnement : dans dix territoires pilotes, des entreprises à but d'emploi (EBE) ont pour charge de recruter en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps choisi tous les demandeurs d'emploi volontaires du territoire au chômage depuis plus d'un an. Les entreprises doivent, dans ce cadre, développer des activités économiques non concurrentes de celles qui sont déjà présentes sur le territoire. Depuis le lancement de l'expérimentation, un emploi a ainsi été trouvé à 900 personnes qui en étaient privées durablement. Le dispositif devait démontrer que son coût ne dépasserait pas la dépense directe et indirecte de la collectivité liée à la prise en charge du chômage de longue durée. S'il est un peu tôt pour évaluer avec précision le gain ainsi généré pour les finances publiques, les premières évaluations parviennent à un montant de près de 14 000 euros par ETP. Surtout, d'un point de vue plus qualitatif, le fait d'inclure dans l'emploi des chômeurs de longue durée non par des contrats précaires ou aidés, mais bien par des CDI, génère une dynamique très positive pour leur parcours de vie comme pour leur territoire. Le tissu associatif se trouve renforcé, de même que l'économie locale, qui bénéficie de leur pouvoir d'achat accru. Dans un souci de transition écologique,

L'heure est à l'accélération du calendrier législatif. Le dernier rapport du comité scientifique d'évaluation confirme qu'une extension de l'expérimentation est désormais envisageable.

l'amélioration de la situation de l'emploi en France demeure fragile et les comparaisons européennes donnent l'impression que nous luttons contre le chômage comme si nous connaissions le plein emploi.

qui doivent constituer un tremplin vers l'emploi de droit commun. À cet égard, je ne peux que m'étonner de la poursuite de l'expérimentation des emplois francs. Plutôt que de nous remettre l'évaluation prévue par la loi de finances pour 2018, vous avez, madame la ministre, décidé de prolonger et de généraliser ce dispositif par décret. Cette méthode ne me semble pas satisfaisante. Au demeurant, force est de constater que le nombre de contrats signés demeure très loin des objectifs que vous vous étiez

même s'il s'agit d'une idée du Président de la République- tout le monde peut se tromper. Aujourd'hui, il serait nécessaire de trouver d'autres moyens de lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qui doit, selon moi, passer par la formation et non par la subvention. J'espère qu'une réflexion plus poussée sera menée lorsque vous déciderez des suites à donner à l'expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée, qui, contrairement aux emplois francs, a fait l'objet d'évaluations publiques. Ces évaluations montrent que, en l'état, un tel dispositif ne peut pas raisonnablement constituer une réponse de grande échelle au chômage de longue durée, malgré les effets positifs qui peuvent être constatés localement. Le plan d'investissement dans les compétences constitue, lui, sur le papier, une réponse plus intéressante. Toutefois, je relève que ce plan comprend, d'une part, des dispositifs pérennes mis en place au cours du quinquennat précédent, et, d'autre part, une enveloppe dont l'utilisation est très peu documentée. Je note d'ailleurs que, pour la deuxième année consécutive, les crédits dédiés au PIC au titre du programme 103 vont finalement baisser. Malgré ces incohérences dans la politique gouvernementale en faveur de l'emploi, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission pour 2020 et des articles qui lui sont rattachés, sous réserve de l'adoption de ses amendements.

Nous constatons que les crédits de paiement de la mission sont maintenus cette année à hauteur de 12,7 milliards d'euros, avec même une légère hausse de 2,58 %. Dans le détail, cela donne deux programmes en hausse et deux programmes en baisse. D'abord, le programme 102, « Accès et retour à l'emploi », et le programme 155, « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail voient leurs crédits de paiement baisser. Le programme 102 baisse de 1,57 %. Malgré la hausse de 1,75 % des crédits alloués à l'action Plan d'investissement des compétences, les deux autres actions du programme emportent une baisse globale de celui-ci.

Notons une baisse de 5,77 % des crédits dédiés à l'action Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et de retour à l'emploi. Cela interroge Ensuite, le programme 103, « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », et le programme 111, « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail », voient leurs crédits de paiement revus à la hausse. Le programme 103 progresse de 8 %. Cette progression est principalement portée par les revalorisations de l'action Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences, ainsi que de l'action Plan d'investissement des compétences. Toutefois, cela se fait au détriment de l'action Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi, qui baisse de 24 %. Cette réduction d'un quart de ce budget est inquiétante. Le programme 111 progresse de 13 % en raison de la réévaluation de 36 % de l'action Dialogue social et démocratie sociale. Cela sera bénéfique. Nous espérons toutefois que ce sera de nature à compenser la baisse de 18 % des crédits alloués à l'action Qualité

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé l'accompagnement de l'apprentissage en France : les régions ne financent plus les et le canal de financement passant par le compte d'affectation spéciale « Financement de la modernisation et du développement de l'apprentissage » (CAS FNDMA) n'a plus lieu d'être. En effet, jusqu'en 2019, une fraction de 51 % du produit de la taxe d'apprentissage versée par les entreprises transitait par le CAS FNDMA et était redistribuée aux conseils régionaux sous forme de « ressource régionale pour l'apprentissage ». L'ensemble de la taxe d'apprentissage sera désormais affectée à France compétences et aux opérateurs de compétences, qui financeront les CFA sur la base d'un financement « au contrat Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit donc la suppression du CAS FNDMA. Par ailleurs, l'État avait mis en place plusieurs dispositifs d'aide à destination des apprentis et de leurs employeurs, ces aides pouvant prendre la forme d'aides directes, d'exonérations d'impôt ou de cotisations sociales et être financées par des crédits budgétaires ou par d'autres moyens- ressources fiscales affectées, dépense fiscale. À compter du 1 janvier 2019, la loi a prévu le remplacement des quatre dispositifs d'aide aux employeurs d'apprentis par la nouvelle aide unique calculée dans le projet de loi de finances pour 2020 pour un montant de 662 millions d'euros. Celle-ci remplace des aides auparavant financées par les régions, ce qui explique l'augmentation de ce budget. Concernant la compétence apprentissage, un financement complémentaire d'un montant de 218 millions d'euros sera versé aux régions en compensation de son transfert.

Les régions seront également destinataires de deux enveloppes distinctes pour financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement des CFA. Je me permets toutefois de rappeler que l'ensemble de ces mesures d'accompagnement financier est jugé insuffisant par Régions de France, qui attendait 369 millions d'euros pour assurer la neutralité financière de la réforme de l'apprentissage et près de 250 millions d'euros pour participer au financement des CFA les plus fragiles. De plus, il pourrait être intéressant que les enveloppes soient sanctuarisées de manière pluriannuelle pour que les régions gardent de la visibilité à moyen et long termes, qu'elles puissent ainsi maintenir des politiques fortes et cohérentes en matière d'apprentissage. Les ressources dédiées à l'apprentissage, sous réserve des décisions du conseil d'administration de France compétences, pourraient s'élever à 5 milliards d'euros. Il convient de préciser que l'affectation des montants par dispositif se fait au terme d'une délibération annuelle du conseil d'administration dans les limites d'une fourchette réglementaire. Cette prévision englobe l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, le financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des régions, ainsi que la péréquation. Actuellement, les régions n'échangent pas sereinement avec France compétences. Il est toujours difficile d'obtenir une information, malgré la présence d'un représentant de l'association Régions de France au sein du conseil d'administration. La transition est donc compliquée par l'absence d'instance de dialogue. Au-delà des calculs de compensation budgétaire, l'État devrait organiser les échanges afin de faciliter le transfert de la compétence apprentissage. En espérant que ces points de vigilance concernant l'apprentissage auront retenu votre attention, le groupe Union Centriste votera, comme le proposent nos rapporteurs spéciaux et notre rapporteur pour avis, les crédits de cette mission. La parole

semble enfin stabiliser ses crédits à leur niveau de l'année dernière. Les autorisations d'engagement s'élèveront ainsi à 13,52 milliards d'euros et les crédits de paiement à 12,78 milliards d'euros pour l'année prochaine. Un soulagement peut-être, mais de courte durée. En effet, les crédits consacrés à l'action de l'État en faveur du travail et de l'emploi restent inférieurs de 2,6 milliards d'euros à ceux de 2018. Lorsque l'on analyse la situation du marché de l'emploi aujourd'hui en France, c'est d'autant plus inquiétant. Le contexte actuel témoigne d'une forme de chômage paradoxale.

Une tendance dont l'équilibre reste déjà précaire. Ces indicateurs masquent une triste réalité : ils gomment les fortes disparités qui fracturent notre territoire, la précarisation de l'emploi et l'éloignement toujours plus important des chômeurs les plus fragiles. En effet, derrière le taux de chômage le plus bas enregistré depuis juillet 2018 par l'Insee se cachent le recul du taux d'emploi à temps complet et la diminution des taux d'emploi et d'activité des jeunes. Pour les publics les plus éloignés de l'emploi, l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) semble avoir tenu ses promesses. Les trois rapports qui vous ont été remis le mois dernier, madame la ministre, concluent à un bilan positif sur les dix territoires tests. L'augmentation de 6 millions d'euros des crédits pour ce dispositif est donc la bienvenue. Mais la question qui se pose aujourd'hui porte avant tout sur l'extension des TZCLD.

Si la mission « Travail et emploi » permet aussi de conforter le grand plan d'investissement dans les compétences lancé par le Gouvernement, les maisons de l'emploi restent, cette année encore, mises à l'écart de la politique de lutte contre le chômage des plus jeunes. Pourtant, les missions locales chargées de la mise en oeuvre de la garantie jeunes partagent l'objectif du PIC d'agir en faveur de la formation et de l'accompagnement de 2 millions de jeunes de 18 à 25 ans d'ici à 2022. Ce plan était attendu et constituait une véritable opportunité pour les acteurs de l'emploi. Néanmoins, il semble être arrivé trop tardivement. Comment armer ces jeunes pour satisfaire aux nouvelles exigences du monde du travail alors que les pratiques des entreprises, dans leur façon de détecter et de recruter, évoluent continuellement ? On observe déjà un basculement de la « recherche de compétences » vers la « recherche de potentiels » des employeurs. Dans ce contexte, les maisons de l'emploi constituent des outils souples et simples qui peuvent être mobilisés rapidement, efficacement, et ce de manière innovante aux fins de répondre aux besoins sans cesse renouvelés du marché de l'emploi. Ces maisons de l'emploi permettent de garantir un socle de services universels de proximité et de remédier aux « angles morts » des politiques publiques. Car le combat contre le chômage et la précarisation du travail ne peut être mené exclusivement par l'État ; ces politiques territoriales et déjà orchestrées dans les métropoles comme en milieu rural, où les élus locaux agissent, sur le terrain, en faveur de l'emploi et des compétences. Le PIC ne saurait atteindre les objectifs qui lui sont fixés sans les fers de lance que représentent ces plateformes locales d'animation et d'ingénierie que sont les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) et les maisons de l'emploi (MDE). La pertinence de ces outils en termes de plan de formation, d'analyse des besoins des entreprises et de gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, ce sont 83 maisons de l'emploi portées par 3 811 communes avec au total de plus 6 millions d'habitants concernés ; ce sont 147 PLIE au service de 5 740 communes qui ont accompagné l'an dernier 130 000 personnes très éloignées de l'emploi, dont 48 % ont trouvé un emploi durable ; ce sont 448 facilitateurs de la clause sociale d'insertion, pour la plupart formés par le réseau Alliance Villes et qui ont développé plus de 15 millions d'heures d'insertion en 2018, soit 38 000 personnes recrutées, dont 53 % l'ont été dans un emploi durable ou en formation au bout de six mois. Il faut soutenir les maisons de l'emploi, qui n'ont toujours pas de programme dédié. Alors que 82 millions d'euros étaient affectés par l'État à ce dispositif en 2010, ce chiffre tombera encore une fois à 5 millions d'euros en 2020, laissant les collectivités en assumer, quasi seules, le financement. C'est pourquoi je remercie le Sénat de se mobiliser de nouveau pour garantir le maintien de ces structures, en les dotant de 10 millions d'euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, et j'espère que le Gouvernement entendra cet appel. Par conséquent, la grande majorité des membres du groupe du RDSE votera, avec la commission des finances, pour l'adoption des crédits de la mission « Travail et emploi », sous réserve de l'adoption de l'amendement des rapporteurs spéciaux relatif aux maisons de l'emploi.

les entreprises n'ont plus peur d'embaucher et elles créent de l'emploi. Les ordonnances Travail leur ont donné un cadre clair, qui permet cette émancipation. Résultat : le taux de chômage est passé de 9,6 % à 8,5 %. Si la réduction du nombre de chômeurs reste la priorité, cette mission s'inscrit dans un projet plus large. Elle instaure une nouvelle politique d'emploi fondée sur les compétences, la liberté donnée aux acteurs et les leviers permettant à chacun d'aller vers l'emploi. Pour ce faire, la mission répond à un double objectif : lutter contre un chômage spécifique- celui qui est vécu par 2 millions de personnes, pour moitié des personnes non ou peu qualifiées et pour moitié des jeunes éloignés de l'emploi l'édification d'une société de compétences, qui passe, en amont, par l'anticipation des mutations économiques et, en aval, par la volonté de donner à chacun la possibilité de choisir son avenir professionnel. Tout cela, c'est l'ADN de la loi du 5 septembre Le PLF pour 2020 poursuit les efforts engagés et son architecture financière le démontre bien. Ainsi, le budget pour la mission s'élève, à périmètre constant, à 13,52 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 12,78 milliards d'euros en crédit de paiement. Cette mission Cette mission se subdivise en quatre programmes. Favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des chômeurs de longue durée, des jeunes sans qualification et des travailleurs handicapés, tel est l'objectif du programme 102, qui obtient les moyens de ses ambitions avec 6,4 milliards d'euros en autorisations d'engagement. est construit autour de trois actions, toutes consacrées à la personne en difficulté et aux outils lui permettant de retrouver un emploi. La première, dotée d'un crédit de 3,5 milliards d'euros, est centrée sur l'amélioration et l'efficacité du service public. l'octroi des moyens nécessaires pour une réponse adaptée aux besoins du demandeur d'emploi, à l'instar d'un soutien dans la recherche d'un emploi, de la personnalisation d'un projet professionnel ou encore de l'accès à de nouvelles compétences. La seconde action, dotée de 2,187 milliards d'euros de crédits, est dévolue à l'amélioration des dispositifs en faveur des personnes les plus éloignées du marché. Des outils puissants seront mis en oeuvre dans le cadre du fonds d'inclusion dans l'emploi, comme l'insertion par les contrats aidés ou par l'accélération de l'accompagnement des publics les plus en difficulté. Pour ce faire, l'augmentation des effectifs de Pôle emploi se traduit par une hausse, en 2020, du plafond d'emplois de 950 équivalents temps plein travaillé (ETPT). cette évolution est assortie une réorientation de l'offre d'accompagnement, en phase avec la situation actuelle du marché du travail et de l'emploi. Enfin, avec un crédit de 589 millions d'euros, la troisième action a pour ambition, au travers du plan d'investissement dans les compétences (PIC), d'accompagner en formation, d'ici à 2022, environ 1 million de jeunes et 1 million de personnes éloignées de l'emploi. Accompagner les mutations économiques et le développement de l'emploi, tel est l'objectif du programme 103. Celui-ci, doté de 6,4 milliards d'euros en autorisations d'engagement, enregistre une hausse de 8 % par rapport à 2019. Il est prioritairement fléché vers un soutien des actifs et des entreprises dans leurs éventuelles phases de transition ou leur montée en compétence. Il accompagne les restructurations sur les territoires, stimule l'emploi et la compétitivité et finance les opérateurs nationaux de la formation professionnelle. Rappelons-le, voilà quinze jours, un outil révolutionnaire a été lancé, l'application mobile « Mon compte formation », l'un des moteurs de ce programme. Ce logiciel permet à chaque actif de sécuriser son parcours professionnel, de se préparer à une transition, voire de changer d'orientation. Accessible à tous, soit à plus de 25 millions d'actifs, elle permet de connaître son budget personnel de formation en temps réel, de comparer plus d'une dizaine de milliers de formations, avant de choisir celle qui correspond le mieux à ses attentes. 25 milliards d'euros de formation ont été mis à la disposition des Français cette application. C'est une clé pour réparer l'ascenseur social. Au-delà de cet outil, deux actions essentielles composent le programme 103. La première, dont le bras armé est le soutien aux contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, permet l'insertion dans l'emploi et la reconnaissance des compétences. Cet axe est primordial ; les moyens financiers sont donc en hausse de 36 % par rapport à 2019. La seconde est la montée en puissance du plan d'investissement dans les compétences ; la formation est en effet la pierre angulaire de l'émancipation. Nous devons donner aux jeunes éloignés du marché du travail et aux demandeurs d'emploi peu qualifiés les outils et les moyens de se former, en particulier dans les nouveaux métiers liés à l'écologie ou au numérique. Environ 14 milliards d'euros de crédits y seront consacrés sur le quinquennat. Améliorer la qualité de l'emploi et les relations de travail, tel est l'objectif du programme 111. Les crédits de celui-ci enregistreront l'année prochaine une hausse de 13 % par rapport à cette année. Ce programme vise à améliorer les conditions d'emploi et de travail des salariés du secteur concurrentiel, au moyen de plusieurs leviers : la qualité du droit et sa diffusion, le contrôle de sa mise en oeuvre, le conseil et l'appui au dialogue social. Deux principales actions composent ce programme. première concerne la santé et la sécurité au travail. La prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail sont des facteurs de compétitivité des entreprises. Cela passe par l'information et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Les crédits dédiés à cette action connaissent une hausse de 13 % par rapport à l'année en cours. La deuxième action concerne le dialogue et la démocratie sociale. éléments contribuent à l'amélioration des conditions de travail et à la compétitivité des entreprises. Or la France n'est pas un exemple en matière de dialogue social. Pour accélérer la mise en oeuvre des mesures contenues dans les ordonnances Travail, les crédits sont en augmentation de 36 % en 2020. Ils serviront notamment à financer les projets liés à la mesure de la représentativité patronale et syndicale. Concevoir, gérer et évaluer les politiques de l'emploi et du travail, tels sont les objectifs du programme 155. Celui-ci est doté d'un budget de 668 millions d'euros en autorisations d'engagement, et son action est également orientée vers la gestion du personnel mettant en oeuvre ces politiques de santé et de sécurité au travail, d'amélioration de la qualité et de l'effectivité du droit, de développement du dialogue et de la démocratie sociale. Mes chers collègues, réparer l'ascenseur social, renouer le dialogue, améliorer les conditions de travail, former et anticiper les transitions sont autant de vecteurs qui permettent le retour à l'emploi et l'augmentation de la compétitivité.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la mission « Travail et emploi » est marquée, cette année encore, par des moyens insuffisants ; en effet, la très légère hausse de ses crédits ne suffit pas à compenser les baisses drastiques des dernières années, des baisses de dépenses qui s'inscrivent dans l'objectif de réduction générale des dépenses publiques. Cela dit, les conséquences de cette politique sont lourdes, affectant directement la vie de femmes et d'hommes qui travaillent ou qui recherchent péniblement du travail. personnes demandent simplement à vivre dignement du fruit de leur travail et à bénéficier d'une protection sociale de qualité. Or comment répondre à cette légitime aspiration quand c'est sur elles que pèsent vos réformes, dont l'objectif affiché serait de leur faire gagner du pouvoir d'achat ou de simplifier leurs démarches ? La réalité est tout autre. Votre réforme de l'assurance chômage est, sur ce point, emblématique. La régression des droits des demandeuses et demandeurs d'emploi vous permettra de dégager 4,5 milliards d'euros d'économies, mais à quel prix ? Plus de 1 million de personnes sont frappées de plein fouet par votre réforme ; 850 000 chômeurs verront leurs indemnités baisser de 20 % et 200 000 autres seront privés de toute indemnité. son côté, Pôle emploi subit depuis deux ans des baisses sévères de budget- 50 millions d'euros d'économies en 2018 et 85 millions en 2019 -, et vous maintenez ce cap, avec 137 millions d'euros de subventions en moins pour 2020, dans le cadre du programme 102. Vous soulignez crânement une augmentation des effectifs de Pôle emploi de l'ordre de 1 000 emplois, mais c'est compter sans la suppression de 800 emplois au cours des deux dernières années. Nous ne sommes pas non plus dupes en ce qui concerne votre tour de passe-passe consistant à faire financer une partie de cette augmentation d'effectifs par l'Unédic, dont la contribution pour Pôle emploi augmente. En somme, ce sont les chômeuses et chômeurs qui financent eux-mêmes cette mesure De même, votre argument consistant à dire que la très légère baisse du chômage justifierait la baisse des subventions pour Pôle emploi est tout bonnement fallacieux. D'abord, la baisse du chômage dont vous vous targuez n'efface pas le taux encore trop important de chômage- le nombre d'inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues, dépasse 6 millions. le nombre de chômeurs de longue durée, quant à lui, continue de progresser. Si l'on veut un meilleur accompagnement des demandeuses et demandeurs d'emploi, il faut nécessairement augmenter les moyens du service public de l'emploi, non les réduire. Du côté de l'inspection du travail, c'est encore une véritable hécatombe ! Cette inspection traverse une lourde crise depuis maintenant de nombreuses années. Vous faites le choix non pas de soulager les inspectrices et inspecteurs du travail, mais de réduire toujours plus leurs effectifs et, plus globalement, les moyens de fonctionnement de l'administration du travail. Le programme 155 voit ainsi ses crédits baisser, en 2020, de 20 millions d'euros, soit de 2,96 %. Vous avez annoncé cette année encore un objectif de diminution de 2,5 % par an des effectifs, d'ici à 2022, sachant que 2 000 départs à la retraite sont prévus pour la même période contre seulement 1 000 recrutements. 15 % des sections seront supprimées. À côté de cela, vous demandez aux inspectrices et inspecteurs du travail de multiplier les contrôles en matière de détachement des travailleurs étrangers,

concerne votre politique d'accompagnement vers et dans l'emploi, on observe, comme le souligne le rapporteur spécial, une baisse de 200 millions d'euros pour les parcours emploi compétences, qui relèvent du programme 102, avec des difficultés persistantes pour le secteur associatif, ainsi qu'une diminution de la moitié des contrats aidés depuis le début

le droit des salariés à la formation tout au long de leur vie professionnelle. Nous regrettons également le désengagement progressif de l'État dans les maisons de l'emploi. À cet égard, l'amendement des rapporteurs tendant à augmenter ces crédits de 5 millions d'euros supplémentaires ne saurait nous satisfaire, puisque cette somme viendrait en déduction des crédits du programme 103.

travers d'exonérations de cotisations sociales, qui dépassent 66 milliards d'euros. Si vous cherchez des moyens, allez les prendre là où ils sont ; c'est le coût du capital qui mine notre économie et qui déséquilibre les comptes sociaux,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons ce matin les crédits de la mission « Travail et Emploi » pour l'année 2020.

Il demeure toutefois notablement plus élevé dans les outre-mer. Ainsi, à La Réunion, c'est près d'un actif sur quatre qui est concerné, Pour ce qui concerne la réduction des dépenses publiques, les crédits de paiement devront atteindre près de 13 milliards d'euros l'année prochaine. Si ce montant paraît en légère augmentation par rapport à 2019, c'est surtout parce que les baisses réalisées précédemment étaient importantes. Je crois qu'il faut donner un satisfecit au travail réalisé par le ministère, qui, d'une part, a strictement respecté la programmation triennale 2018-2020 et qui, d'autre part, a contribué de façon significative à l'effort de réduction de la dépense publique. Cette contribution démontre, si besoin en était, qu'on ne redynamise pas le marché du travail en dépensant sans compter. Bien sûr, le fait que le chômage reflue parallèlement à la diminution des dépenses ne prouve pas que la baisse du premier entraîne mécaniquement la baisse des secondes, mais cela démontre à tout le moins que l'un n'empêche pas l'autre. Pour vaincre le mal français, on peut donc aussi se passer de politiques dispendieuses ... Je salue ici le choix qui a été fait de focaliser les politiques sur les publics les plus éloignés de l'emploi. Il s'agit donc non pas de supprimer purement et simplement les moyens soutenant les politiques de cette mission, mais bien d'opter pour une allocation optimisée des ressources ; en la matière, l'efficience est souvent gage d'efficacité. C'est notamment le cas des crédits portant sur l'insertion par l'activité économique. Cela a déjà été rappelé, les montants qui y seront consacrés l'année prochaine devraient dépasser 1 milliard d'euros. Il s'agit de dispositifs éprouvés par le terrain et par les retours d'expérience, sur lesquels nous avons raison de capitaliser. pour le plan d'investissement dans les compétences ; les moyens qui y sont alloués constituent un élément clé pour dépasser le paradoxe, malheureusement très français, de chômeurs qui peinent à retrouver un emploi et d'entrepreneurs qui peinent à recruter des employés. La montée en compétences doit permettre d'ajuster le marché du travail afin que la demande s'adapte mieux à l'offre. Le marché de l'emploi ne saurait pourtant se réduire à un schéma simpliste, avec, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les employés. Le fait de sortir du salariat, par l'initiative individuelle, la création d'entreprise, s'avère parfois plus efficace pour lutter contre le chômage. C'est pourquoi le dispositif de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise a connu un si grand succès en France, notamment auprès des publics éloignés de l'emploi, qui rencontrent le plus de difficultés à s'insérer durablement sur le marché du travail. Le Gouvernement a fait le choix de l'étendre à tous les publics à compter de 2019. Je comprends et partage cette ambition, mais force est de reconnaître que des effets indésirables se sont déjà fait sentir ; c'est pourquoi je pense qu'une application plus rigoureuse est indispensable à la pérennité du dispositif. cette restriction du dispositif ne doit pas remettre en cause les équilibres financiers des entrepreneurs qui se sont lancés dans l'aventure, dans des conditions qu'il s'agirait maintenant de changer, alors qu'ils ont déjà pris un risque. raison pour laquelle je soutiens l'amendement déposé au nom de la commission des finances par notre excellent rapporteur spécial Emmanuel Capus. Très bien ! Un encadrement plus strict, mais surtout plus juste, du dispositif est nécessaire. De même, l'amendement qui vise à augmenter de 5 millions d'euros les crédits alloués aux maisons de l'emploi me semble pertinent. Il s'agit de renforcer ainsi le réseau d'accompagnement à destination des demandeurs d'emploi, afin de faciliter leur insertion durable dans le marché du travail. C'est une mesure vitale pour le dynamisme économique de nos territoires et pour la cohésion sociale de notre pays. Le groupe Les Indépendants votera les crédits de cette mission ainsi amendés.

la France s'est bâtie, rappelons-le, sur un système de gestion paritaire, qui renvoie à une pratique de régulation sociale ; il s'agit, sans doute faut-il le rappeler, d'un point d'équilibre de notre société, dont nous savons combien elle est fragile. Mon intervention portera principalement sur le sujet de l'assurance chômage ainsi que sur le bonus-malus.

Nous vous l'avons dit, madame la ministre, même si nous validons certaines des mesures proposées, il nous semble que le passage en force se paie toujours et que notre pays reste socialement fragile. Ce passage en force se matérialise également dans le financement de Pôle emploi et dans ses effectifs supplémentaires. En effet, si le nombre d'emplois progresse de 1 000 unités sur trois ans, conformément aux annonces de l'été, nous ne pouvons que regretter un paradoxe apparent : l'augmentation affichée des emplois s'accompagne d'une baisse du financement de l'État, la subvention pour charges de service public passant de 1,3 milliard d'euros en 2019 à 1,2 milliard d'euros en 2020, soit une baisse de 10 %. Lors de votre audition, madame la ministre, que ce montant tenait compte de la poursuite des efforts engagés par l'opérateur, mais,, il faut bien considérer que, conformément à ce qu'ont dit mes collègues, ce sont les demandeurs d'emploi indemnisés qui vont compenser cette baisse. effet, en parallèle, la contribution de l'Unédic au financement de Pôle emploi augmentera de 10 % à 11 %, ce qui réduit d'autant les sommes disponibles pour l'indemnisation. Nous ne pouvons que regretter la forme de ces décisions, qui, par un tour de passe-passe du Gouvernement, ont imposé aux employeurs de financer davantage Pôle emploi, tout en baissant ses propres financements. Un mot sur le bonus-malus.

permettant la mise en place de majorations applicables pour les CDDU et les CDD de moins de trois mois, mais la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 avait mis fin à cette modulation, car la surtaxation des contrats courts n'avait pas eu d'impact mesurable sur le recours à ces contrats.

Je me félicite donc du vote de la commission des affaires sociales, qui a supprimé les dispositions de l'article 8 du PLFSS, relatif à ces enjeux de bonus-malus, même si je crains que mon bonheur ne soit que de courte durée

Cela étant, nous veillerons à l'impact du bonus-malus, de sorte que celui-ci ne soit pas,, un impôt complexe à mettre en oeuvre de plus. Quant à Pôle emploi, nous continuons à considérer qu'il est risqué de le rendre encore plus dépendant des ressources de l'assurance chômage ; dans ce pays, le paritarisme ne peut pas se contenter d'incantations

à dire « non »- je l'ai entendu -à la dégradation des services publics, à cette déshumanisation, à la dévitalisation de nos territoires. Plus de 1 million de Français ont manifesté pour exprimer leur désaccord et leur mécontentement ; entendez-les, madame la ministre De même, je ne peux aborder la discussion sur cette mission sans parler de l'assurance chômage. Alors que l'enjeu de la sécurisation des parcours professionnels n'a jamais été aussi important, votre réforme, dont la première phase est entrée en vigueur le 1 novembre dernier,

la moitié des demandeurs d'emploi indemnisés qui travaillent ne seront plus du tout indemnisés ou le seront moins ; c'est ça la réalité ! Votre parti pris est clair : vous supposez que la baisse des allocations incitera les bénéficiaires à trouver plus rapidement un travail. Un tel raisonnement laisse entendre que les chômeurs seraient responsables de leur situation ; cela n'est pas acceptable. Madame la ministre, les allocations ne sont pas des libéralités consenties par le prince ; ce sont des cotisations et des droits réels créés par le travail. Les partenaires sociaux, les associations de lutte contre la pauvreté vous l'ont dit : cette réforme est injuste et brutale ; elle abîme notamment ce qui fut un grand progrès social les droits rechargeables. Ne l'oublions pas, un chômeur sur deux n'est déjà pas indemnisé, 2,6 millions de chômeurs touchent moins de 860 euros par mois 60 % des chômeurs ne vont pas au bout de leurs droits. Voilà qui devrait vous inciter à renoncer à cette réforme ou alors à l'assumer pour ce qu'elle est : une réforme financière, dont vous attendez des milliards d'économies, au détriment des plus fragiles de nos concitoyens.

Ainsi, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit de diminuer de près de 137 millions d'euros la subvention pour charges de service public attribuée à Pôle emploi. Cette réduction s'ajoute à deux précédentes baisses- 50 millions d'euros en 2018 et presque 85 millions d'euros en 2019 -, ce qui traduit le désengagement progressif de l'État dans le financement de Pôle emploi. deviendra encore plus dépendant des ressources de l'assurance chômage, et ce contre l'avis des partenaires sociaux, puisque la contribution de l'Unédic, portée à 11 % de ses ressources, Vous prétendez ainsi renforcer l'accompagnement des chômeurs, dont, je le répète, vous diminuez les allocations, mais force est de constater que ce sont les chômeurs eux-mêmes, au travers d'une nouvelle ponction dans les caisses de l'Unédic,

Vous nous annoncez une augmentation des effectifs de Pôle emploi, mais celle-ci ne sera pas de nature à compenser les baisses, très fortes, enregistrées au cours des dernières années. C'est oublier aussi que cette hausse a surtout vocation à renforcer l'accompagnement des entreprises et non celui des demandeurs d'emploi, des plus éloignés du marché du travail. J'en viens maintenant au plan d'investissement dans les compétences, lequel traduirait, selon le Gouvernement, « à la fois la volonté de miser sur les qualifications, de démontrer que tout n'est pas joué à la fin de la scolarité, de ne laisser personne au bord de la route et de transformer le système de formation pour soutenir la compétitivité des entreprises Dès lors, la diminution de 120 millions d'euros des crédits du PIC constitue un bien mauvais signal. Alors que la formation des chômeurs était affichée comme une priorité, elle se révèle constituer la variable d'ajustement du Gouvernement. C'est difficilement compréhensible.

Les résultats, somme toute modestes, des PEC, dont les crédits ont été sous-consommés en 2018, soulignent l'inadaptation de ce dispositif à une large partie des publics précédemment concernés par les contrats aidés, ainsi qu'à de très nombreuses associations employeurs.

ce montant reste insuffisant. C'est pourquoi notre groupe défendra un amendement visant à porter leurs crédits à 10 millions d'euros. Pour terminer, j'évoquerai l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée », que je connais bien. À Colombelles, dans mon département du Calvados, l'expérience menée est très positive et concluante, de sorte que je suis favorable à son extension. C'est d'ailleurs ce qu'avait promis le Président de la République, voilà déjà plus d'un an, à l'occasion de la présentation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. J'y reviendrai, là aussi, par voie d'amendement, en insistant sur la dimension sociale et humaine du dispositif. Madame la ministre, la diminution des effectifs de votre propre ministère, dont ceux de l'inspection du travail, constitue en elle-même un très mauvais signal, à une époque marquée par des modifications substantielles du droit du travail et alors que la lutte contre le travail illégal doit tous nous préoccuper. Vous avez, par ailleurs, acté, sans explication, la disparition du Haut Conseil du dialogue social dans une annexe budgétaire au présent projet de loi de finances, au motif de sa redondance supposée avec la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il n'est jamais souhaitable de supprimer une instance sans concertation ni évaluation préalable, surtout lorsqu'elle oeuvre au dialogue social. J'y reviendrai dans quelques instants. instants. Pour toutes les raisons évoquées, les sénateurs du groupe socialiste et républicain prendront leurs responsabilités, en ne votant pas les crédits de la mission « Travail et emploi ». La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme à l'accoutumée, l'examen annuel des crédits de la mission « Travail et emploi » est l'occasion pour moi d'évoquer la situation des maisons de l'emploi et de la formation. J'ai choisi de concentrer mon propos, dans un premier temps, sur la question des missions locales et des maisons de l'emploi, dont je connais l'action, notamment sur mon territoire de l'Aisne, depuis 1995. Alors que la dotation s'élevait encore à 11,5 millions d'euros en 2018, l'engagement de l'État dans les maisons de l'emploi et de la formation a été divisé par deux, pour tomber à 5 millions d'euros en 2019. La volonté des pouvoirs publics étant de supprimer totalement l'investissement dans ces structures, ce sont par conséquent les collectivités qui les soutiennent financièrement, à bout de bras, avec le concours du Fonds social européen. Amorcer la suppression des maisons de l'emploi est une véritable erreur politique de la part du Gouvernement, alors même que le Président de la République a annoncé son engagement de multiplier par cinq l'accompagnement des jeunes dans le plan Pauvreté.

sont d'autres éléments qui contredisent totalement cette promesse gouvernementale. En outre, elles n'augurent rien de bon pour la lutte contre le chômage de longue durée et la difficulté d'insertion des jeunes et des personnes handicapées sur le marché du travail. utilisée dans un article de l'édition du journal parue hier, c'est un véritable et « vaste plan social » contre les publics précaires et fragiles que le Gouvernement s'attelle à mettre en oeuvre depuis deux ans. Sous couvert de remédier à d'hypothétiques pratiques abusives, le ministère a divisé sa contribution financière dans les contrats aidés par deux. Enfin, en réduisant leur durée maximale de dix-huit à huit mois et de 35 à 20 heures hebdomadaires, vous avez confirmé, madame la ministre, que vous alimentiez vous-même la précarité que vous prétendez tant combattre, en y envoyant obstinément tout un segment démuni de la population. Vous avez justifié, avec cette même philosophie, la baisse des dotations des maisons de l'emploi et de la formation, invoquant la baisse du taux de chômage, passé sous la barre des 9 % au quatrième trimestre de 2018, et la reprise par Pôle emploi de leurs activités. Vous omettez toutefois de préciser, délibérément ou non, que le taux de chômage est en hausse constante chez les catégories B et C et que Pôle emploi ne saurait assurer le même accompagnement des publics jeunes que celui que fournissent les maisons de l'emploi et de la formation Les MEF ont prouvé à maintes reprises leur rôle déterminant dans l'exercice d'un service public de proximité permettant l'accompagnement vers l'emploi et l'insertion des publics vulnérables. Leur assise de proximité les dote d'une capacité à identifier des publics invisibles, condamnés à rester hors des radars d'une aussi grande structure que Pôle emploi, à savoir les jeunes de 16 à 18 ans ou d'échec dans celui-ci, les 26 à 30 ans bénéficiaires du RSA, les moins de 26 ans sans qualification, sans solution d'apprentissage ou avec une solution inadaptée à leurs compétences et leurs aspirations, voire les jeunes frappés d'illettrisme. de la formation occupent une place de premier choix, indispensable dans le tissage de réseaux, grâce à leurs moyens de mobilisation et de concertation, mais aussi à leur capacité à concourir au développement de projets locaux. 60 % des jeunes passés par ces structures sortent avec une qualification ou un emploi et 72 % signent un CDI après dix-huit mois de contrat. Leur efficacité n'est plus à prouver.

La maison de l'emploi et de la formation de Laon, qui a été créée en 2007, travaille depuis deux ans en concertation avec un large panel d'acteurs institutionnels et un réseau de soixante entreprises intégratrices prêtes à accueillir des étudiants en alternance pour mettre en place une école de la seconde chance. Or toutes Or toutes les démarches engagées pour défendre ce projet se heurtent au silence de l'État. Aucune réponse positive n'a été donnée à l'appel à projets lancé par la Direccte, alors même que notre nouveau préfet vient de s'engager à faire de la lutte contre l'illettrisme la première de ses priorités. Je viens d'ailleurs de vous adresser un courrier à ce sujet, madame la ministre, pour obtenir des réponses. Pourquoi l'État ne prend-il pas davantage en compte le travail de terrain et fuit-il le dialogue sur le sujet ? Il est de sa responsabilité de soutenir les initiatives des maisons de l'emploi et de la formation et de reconnaître leur rôle déterminant dans la délivrance d'un service de proximité, notamment auprès des jeunes publics. C'est pour l'ensemble de ces raisons que je soutiendrai l'amendement des rapporteurs spéciaux Emmanuel Capus et Sophie Taillé-Polian, ainsi que celui de mon collègue Michel Forissier en faveur du maintien d'un financement par l'État des maisons de l'emploi et de la formation à hauteur de 5 millions d'euros. S'ils sont adoptés, je voterai les crédits de la mission « Travail et emploi ». Très bien

Je suis ravie de vous retrouver après mon audition du 20 novembre dernier pour poursuivre nos échanges et répondre à vos questions sur la mission « Travail et emploi » du projet de loi de finances pour 2020.

sur les compétences et la liberté donnée aux acteurs : les ordonnances Travail, l'apprentissage, la formation- notamment le plan d'investissement dans les compétences et « Mon compte formation » -, l'assurance chômage. Notre conviction est très claire : la clé de voûte de notre politique, c'est à la fois la lutte contre le chômage et l'émancipation de chacun par la compétence et l'évolution du travail.

À cet égard, 2020 doit être l'année de consolidation et d'approfondissement de la mise en oeuvre opérationnelle de ces transformations, notamment de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

en crédits de paiement. Il est stable en autorisations d'engagement, et il progresse de 210 millions d'euros en crédits de paiement, ce qui montre notre volonté de poursuivre les efforts de transformation.

stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Pendant plus de six mois, nous avons mené une concertation avec les représentants du secteur, dont le résultat a été présenté au Président de la République le 10 septembre dernier à Bonneuil-sur-Marne et a abouti à un « pacte d'ambition pour l'IAE

puissent accéder à l'insertion par l'activité économique dès 2020. Pour cela, le budget est augmenté de 120 millions d'euros, dépassant, pour la première fois de notre histoire, la barre symbolique du milliard d'euros.

L'appui financier de l'État se poursuit en 2020 sur ce sujet, avec un budget de 403 millions d'euros, en augmentation de 7 millions d'euros. Grâce à ce budget et à la contribution de l'Agefiph, ce sont près de 10 000 personnes supplémentaires qui pourront accéder aux entreprises adaptées

en progression de 6 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2019. L'effort supplémentaire de l'État s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et permettra la montée en charge du dispositif dans les territoires qui participent à l'expérimentation, conformément à la loi de 2016, avec 1 750 ETP financés l'année prochaine, contre 811 actuellement embauchés. Je rappelle que le ministère du travail est le principal et parfois l'unique financeur de cette expérimentation, avec une

Cette expérimentation est intéressante. Elle permet de tester des modalités innovantes et très mobilisatrices sur le terrain de lutte contre le chômage de longue durée. L'approche territoriale et la mobilisation des élus locaux constituent notamment un élément essentiel du dispositif.

La hausse de leurs crédits s'établira à 21 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2019, pour un montant total de 371,94 millions d'euros.

Ce montant intègre aussi le financement de la mise en oeuvre de l'obligation de formation instaurée par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, qui est en phase de lancement expérimental.

un meilleur accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises, la responsabilisation des employeurs quant à la précarité des contrats et l'adaptation des indemnisations au contexte actuel.

dans ce budget et dans les décisions de France compétences, de compenser à la fois la perte de la compétence apprentissage, pour les régions

: La parole est à Mme Corinne Féret. La situation de l'emploi est fragile et certaines catégories de personnes demandeuses d'emploi restent très éloignées du marché du travail. Ce sont elles que nous avons le plus de mal à toucher, dans un contexte à la fois de baisse de moyens- je pense en particulier à Pôle emploi -et de fort développement des emplois précaires. À cet égard, je souhaite y insister, la politique de casse des emplois aidés a été dramatique pour ces publics,

De plus, les PEC ne couvrent pas les mêmes publics. C'est pourquoi nous relayons la demande du secteur associatif de créer un nouveau dispositif pour des emplois d'utilité citoyenne. Cette mesure, qui viendrait essentiellement en appui de projets associatifs dans les champs éducatif, environnemental, scientifique, social,

Ce dispositif, inspiré de plusieurs expériences de ces dernières décennies et en tirant les leçons, dote les emplois d'utilité citoyenne d'une aide sur trois ans maximum, dont l'attribution serait fonction de critères d'intérêt général et qui représenterait de 40 % à 80 % du SMIC. L'association employeur devrait démontrer sa capacité à présenter et à gérer un projet d'activité, à analyser et à répondre à des besoins non ou insuffisamment satisfaits ayant un impact social sur la population de son territoire, à mobiliser les acteurs et à développer les partenariats financiers, à présenter un plan de développement pluriannuel incluant les formations éventuellement nécessaires à la qualification des emplois. Cette aide serait versée par l'intermédiaire d'un fonds au sein du budget de la mission « Travail et emploi ». Nous proposons de financer ces emplois par les enveloppes non consommées des PEC, soit 200 millions d'euros.

pour les personnes concernées- je pense notamment aux réductions de la protection chômage qui viennent d'entrer en application. Le plan d'investissement dans les compétences n'échappe pas à cette constatation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

par l'ensemble des interlocuteurs et partenaires. Comme l'année dernière, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à permettre le maintien d'une ligne de crédit à hauteur de 5 millions d'euros, sur proposition de la rapporteure spéciale. Comme l'année dernière, notre analyse de leurs besoins nous porte à juger ce montant insuffisant, au risque d'un saupoudrage peu efficace ou d'une fermeture

notamment en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur les clauses sociales. Les maisons de l'emploi peuvent jouer un rôle d'ingénierie important

aux deux années suivantes. En 2019, conformément aux promesses de campagne d'Emmanuel Macron, ce dispositif est devenu l'ACRE et a été étendu à tous les créateurs ou repreneurs d'entreprise.

Quoi qu'il en soit, les personnes concernées ont vraisemblablement compté sur cette aide dans leur plan d'affaires, aux taux initialement prévus. Il est donc vraiment regrettable que l'État revienne sur sa parole. C'est également juridiquement risqué, puisque c'est contraire, selon nous, au principe d'espérance légitime.

Partant de ce principe, qui est faux- c'est un sophisme que vous avez établi -, vous avez puni tous les chômeurs. Ainsi, 1,3 million d'entre eux vont se trouver en difficulté. Certains ne toucheront même plus d'allocations chômage. Leur famille, leurs enfants vont en pâtir.

du Haut Conseil du dialogue social et des défenseurs syndicaux. Vous avez déjà été interpellée sur le sujet, madame la ministre, puisque cet amendement reprend celui du rapporteur pour avis de l'Assemblée nationale. Ce dernier relevait la suppression du Haut Conseil dans l'annexe budgétaire au projet listes des commissions, instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, sans que celles-ci soient parallèlement inscrites dans le projet annuel de performance de la mission « Travail Travail et emploi ». Sur quelle évaluation se fonde donc cette disparition, apparemment programmée ? Je vous ai moi-même interrogée lors de votre audition devant la commission des affaires sociales, mais je n'ai pas été convaincue par votre réponse. Vous avez affirmé qu'il s'agissait de fusion et que les missions du Haut Conseil du dialogue social seraient reprises intégralement. Notre amendement a donc pour objet une évaluation globale du Haut Conseil, afin de permettre au Parlement d'apprécier si cette fusion peut se justifier du fait de sa redondance supposée avec la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et de jouer pleinement son rôle de contrôle, en s'assurant de la reprise effective et de la pérennité des missions concernées dans ce transfert.